L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, présentée par MM. Hervé Maurey et Louis Nègre

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le quatrième paquet ferroviaire, adopté en décembre 2016, a fixé des échéances très claires pour l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs : le 3 décembre 2019 pour les services conventionnés, TER et TET ; le 14 décembre 2020 pour les services librement organisés, c'est-à-dire les TGV, avec une obligation de transposition de la directive d'ici au 25 décembre 2018. Les échéances sont donc proches et l'expérience de la libéralisation du fret ferroviaire nous montre qu'il faut anticiper cette réforme le plus en amont possible. C'est pour cela, mais aussi parce que nous pensons, Louis Nègre et moi-même, que l'ouverture à la concurrence peut et doit être une chance pour le secteur ferroviaire en général, la SNCF en particulier et surtout pour les usagers, que nous avons décidé de travailler à la rédaction d'une proposition de loi dès le début de l'année 2017. Qu'il me soit, à ce stade, permis de saluer le travail et l'engagement constant sur cette question de notre ancien collègue Louis Nègre,

Nous savions que l'ancien gouvernement ne se saisirait pas de ce dossier avant les échéances électorales et nous nous doutions que le gouvernement issu des élections du printemps aurait certainement d'autres urgences. Nous avons donc préparé cette proposition de loi en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes : syndicats, usagers, régions, ARAFER, groupe public ferroviaire, nouveaux entrants et, bien sûr, ministères. Dès votre nomination, madame la ministre, nous vous avons fait part de notre initiative, en vous indiquant que notre démarche visait non pas à gêner le Gouvernement, encore moins à le court-circuiter, mais, au contraire, à mettre à sa disposition notre travail, pour qu'il s'en saisisse le plus rapidement possible. Nous n'avons d'ailleurs pas manqué de vous alerter sur la nécessité de légiférer rapidement, pour définir les modalités de cette réforme d'ampleur. Nous avons déposé notre texte le 6 septembre 2017 et nous vous l'avons présenté dans l'esprit de coconstruction qui était le nôtre. À votre demande, j'ai accepté de renoncer à l'inscription de ce texte à l'ordre du jour en janvier, comme cela était prévu, car vous souhaitiez attendre les conclusions de la mission de M. Spinetta. J'ai accédé à votre souhait, car vous m'aviez assuré que cette proposition de loi serait le véhicule législatif soutenu par le Gouvernement pour mener à bien sa réforme. Profitant de ce délai supplémentaire pour conforter la qualité juridique du texte, le président du Sénat a saisi le Conseil d'État, comme la Constitution le lui Celui-ci a rendu son avis le 22 février dernier. Je tiens à souligner le caractère tout à fait exceptionnel de cette démarche, puisque seules quatre propositions de loi d'initiative sénatoriale avaient été précédemment soumises au Conseil d'État. Quelle ne fut donc pas notre surprise d'apprendre que le Gouvernement décidait finalement de procéder à la réforme du système ferroviaire par ordonnances ! Comment ne pas y voir un mépris absolu du travail du Sénat, du Parlement dans son ensemble et, au-delà, de nos compatriotes, car, sur un tel sujet, un vrai débat s'impose ? La raison invoquée par le Gouvernement est qu'il faut aller vite. Tout à fait d'accord, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de lancer les concertations ? Vous saviez, madame la ministre, que ces échéances existaient ; Louis Nègre et moi-même vous les avions rappelées à plusieurs reprises. Le Gouvernement a préféré prendre son temps, pour ne pas dire le perdre. Aujourd'hui, la concertation avec les syndicats est une priorité, mais pourquoi, au nom de cette concertation, refuser le débat avec le Parlement ? Le Gouvernement ne serait-il pas plus fort s'il pouvait s'appuyer sur un soutien du Parlement ? J'observe d'ailleurs avec étonnement que vous avez, depuis l'origine, voulu éluder le débat sur le sujet. Le transport ferroviaire a été écarté des Assises nationales de la mobilité, au motif qu'un expert aux compétences reconnues dans le secteur aérien allait nous expliquer comment sauver le secteur ferroviaire. L'avenir du système ferroviaire concerne tout de même, vous le savez mieux que quiconque, 3,2 millions de voyageurs par jour. Pourquoi avoir sacrifié le nécessaire débat, dans l'attente des oracles de M. Spinetta, devenu, en quelque sorte, le « gourou » du ferroviaire ? ? Aujourd'hui, pour justifier les ordonnances, vous invoquez, après avoir perdu beaucoup de temps, la nécessité d'aller vite. Mais savez-vous, madame la ministre, qu'il faut en moyenne six mois pour examiner un projet de loi en procédure accélérée, alors que le délai moyen entre la demande d'habilitation par le Parlement et la signature de l'ordonnance est de dix-huit mois ? Ce n'est pas moi qui le dis, mais les statistiques qui l'attestent. En l'espèce, nous avons, vous avez, une proposition de loi qui est prête, qui a été examinée par le Conseil d'État qui, à la suite de cet avis du Conseil d'État, a été améliorée grâce au travail de notre rapporteur en commission. Vous avez donc, grâce à ce texte, la possibilité d'aller plus vite que par ordonnances, lesquelles, dans le meilleur des cas, ne seraient pas adoptées avant le mois de juin. En même temps, vous avez la possibilité de permettre un vrai débat parlementaire. Madame la ministre, jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été décidée par ordonnances, en demandant des habilitations aussi floues. floues. Vous allez nous répondre qu'au fur et à mesure de l'examen de la loi d'habilitation vous introduirez des dispositions législatives définitives. Cette démarche pour le moins inédite, pour ne pas dire exotique, n'est pas de nature à nous rassurer,

Il y a également fort à parier que le Parlement sera, comme c'est souvent le cas, saisi tardivement et aura, de ce fait, peu de temps pour les examiner et mener les concertations nécessaires. L'expérience nous montre en effet que le Gouvernement nous saisit trop souvent au dernier moment de ses amendements, parfois même quelques heures avant l'ouverture de la séance. Je voudrais, avant de conclure, évoquer deux points fondamentaux pour nous. Premièrement, l'ouverture à la concurrence doit se traduire non pas par une dégradation de la qualité du service offert aux clients, mais par une amélioration. Deuxièmement, l'ouverture à la concurrence ne doit pas se faire au détriment des territoires. Nous sommes donc en désaccord total avec la position de M. Spinetta, préconisant de recentrer le ferroviaire sur « les dessertes à grande vitesse entre les principales métropoles françaises Cette position est en contradiction absolue avec le concept d'aménagement du territoire, auquel nous sommes particulièrement attachés. De même, nous ne sommes pas favorables à une ouverture à la concurrence des services TGV reposant exclusivement sur le libre accès au réseau, ce que l'on appelle l', car car elle aboutirait à la disparition de nombreuses liaisons, moins rentables ou déficitaires, mais pourtant indispensables à l'aménagement du territoire. Nous voulons éviter un tel écrémage, du type de celui qui est opéré par les opérateurs de téléphonie, et préserver la desserte des villes moyennes par les services TGV. ce texte, nous proposons donc une mesure forte, pour répondre à la nécessité de préserver l'aménagement du territoire, en prévoyant que l'État, en tant qu'autorité organisatrice de transport, conclura des contrats de service public pour les services TGV,

Madame la ministre, vous l'avez compris, nous sommes favorables à une réforme ambitieuse du système ferroviaire et de la SNCF, ainsi qu'à son ouverture à la concurrence, mais pas dans ces conditions. Grâce à cette proposition de loi, le débat que le Gouvernement voulait nous refuser aura lieu. Je remercie chaleureusement tous les groupes du Sénat qui ont souhaité ou accepté son inscription à l'ordre du jour de notre assemblée. Nous ne sommes pas, sur ces travées, tous d'accord sur le texte que je présente ce soir. Mais nous avons tous la volonté que le débat ait lieu. Nous sommes tous attachés à sauver le système ferroviaire et la SNCF. Nous voulons tous éviter que cela se fasse au détriment de la qualité du service et de la desserte équilibrée de nos territoires. C'est là tout l'enjeu de ce débat. Ces points essentiels constituent le socle commun aux membres de notre Haute Assemblée, dont vous mesurerez ce soir, une fois encore, l'engagement sur ces sujets. La parole

rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ah ! Comme le président Maurey, je m'interroge : pourquoi avoir tant tardé à s'emparer du sujet de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs Ce retard nous oblige, à quelques mois de la date butoir fixée par l'Union européenne, à légiférer par voie d'ordonnances, contribuant à nous priver d'un débat pourtant indispensable. L'ouverture à la concurrence est une obligation européenne. Nous pouvons la transformer en opportunité pour nos transports ferroviaires, qui ont perdu de leur attractivité ces dernières années. Depuis 2011, la fréquentation des trains recule, alors que celle des autres modes de transport- voiture particulière, avion, autocar -progresse. Cette évolution va à l'encontre du modèle que nous devrions défendre pour protéger l'environnement. Elle est à l'opposé de ce qui s'observe chez nos voisins européens, où la part modale du train progresse. Nombre d'entre eux n'ont d'ailleurs pas attendu le quatrième paquet ferroviaire pour ouvrir leurs services à la concurrence, avec des effets positifs sur la qualité de service, sur la fréquentation, sur la réduction des coûts, au profit, bien entendu, des usagers. C'est la raison pour laquelle nous soutenons, sur le fond, cette réforme, à la condition d'en définir correctement les modalités. Tel est l'objet de cette proposition de loi. Nous nous sommes d'ailleurs attachés, en commission, à clarifier et sécuriser plusieurs dispositions du texte sur le plan juridique, en prenant en compte les observations formulées par le Conseil d'État. C'était l'objectif de cette saisine. Comme l'a indiqué le président Maurey, l'un des axes forts de la proposition de loi est de chercher à préserver les dessertes TGV considérées comme peu rentables ou même déficitaires, alors qu'une ouverture à la concurrence reposant exclusivement sur le libre accès au réseau prévu par l'Union européenne, l', aboutirait à un écrémage des dessertes. Aussi la proposition de loi prévoit-elle que l'État conclura des contrats de service public pour l'exploitation des services dits TGV, en combinant des liaisons rentables et des liaisons non rentables. Il s'agit, à ce jour, de la seule solution permettant de préserver de façon certaine des dessertes considérées comme non rentables dans le contexte de l'ouverture à la concurrence, sans rupture de charge pour les usagers. À l'inverse, un conventionnement des seules liaisons non rentables, notamment celles qui permettent de desservir les villes moyennes par des trains TGV, obligerait les usagers à changer de train pour commencer ou terminer leur trajet, ce qui réduirait ce qui réduirait d'autant l'attractivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport. L'objectif est non pas de couvrir tous les services TGV par des contrats de service public, mais de faire coexister, dans un système équilibré, des services librement organisés, en, et des services conventionnés, comprenant des services à grande vitesse. Il reviendra à l'État, en tant qu'autorité organisatrice, de prendre ses responsabilités dans ce domaine, en déterminant les dessertes qu'il souhaite préserver et en concluant les contrats de service public correspondants. Les autres dispositifs de la proposition de loi visent à lever les obstacles à une ouverture effective à la concurrence. Le premier sujet, primordial, est la question des données, car les autorités organisatrices ne parviennent pas, aujourd'hui, à obtenir de l'opérateur historique les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs missions. Pour y remédier, l'article 7 crée un dispositif contraignant, imposant à SNCF Mobilités et SNCF Réseau de transmettre aux autorités organisatrices les informations indispensables à l'exercice de leur mission, assorti d'une possibilité de sanction par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'ARAFER, en cas de manquement. Les autorités organisatrices devront, quant à elles, fournir aux candidats aux appels d'offres les informations nécessaires à la préparation de leur candidature, comme le prévoit l'article 2. Dans les deux cas, un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'ARAFER, déterminera un socle minimal d'informations à transmettre pour fixer un cadre homogène et éviter que des contestations ne bloquent la transmission de ces données. Le deuxième sujet, c'est celui du transfert de personnels entre entreprises ferroviaires. L'article 8 de la proposition de loi fixe, de manière précise et détaillée, le régime applicable au transfert des salariés, ce qui lui confère une garantie juridique forte et limite les incertitudes qui résulteraient d'un dispositif trop flou. Ce dernier laisserait des marges d'interprétation et, donc, des possibilités de contentieux au moment du transfert. L'article prévoit que le périmètre des salariés à transférer est arrêté par les autorités organisatrices de transport et communiqué aux opérateurs souhaitant candidater aux appels d'offres. Le transfert s'effectuera prioritairement sur la base du volontariat, puis sur décision de l'entreprise ferroviaire sortante si le nombre de volontaires est inférieur au périmètre arrêté par les autorités organisatrices. L'article 8 détermine ensuite le socle de droits sociaux garantis aux salariés de SNCF Mobilités transférés, ce que l'on appelle parfois le « sac à dos social » : l'ensemble des salariés conserveront un niveau de rémunération identique à celui qui aura été perçu lors des douze derniers mois précédant le transfert, ainsi que le bénéfice des facilités de circulation en outre, les salariés sous statut garderont leur affiliation au régime spécial de retraite de la SNCF et les droits à pension qui en découlent, ainsi que la garantie de l'emploi. À l'issue d'un premier transfert, les salariés qui seraient amenés à rejoindre de nouveau SNCF Mobilités pourront réintégrer le statut s'ils en bénéficiaient initialement. S'ils sont transférés à un nouvel opérateur, leurs droits garantis seront maintenus. En ce qui concerne les matériels roulants, les autorités organisatrices seront libres de déterminer l'option la plus adaptée elles pourront avoir recours à une société de location, demander aux entreprises d'apporter leurs propres matériels, ou récupérer la propriété des matériels de SNCF Mobilités pour les mettre à la disposition de l'entreprise remportant le marché. De la même façon, en vue de faciliter l'accès des entreprises ferroviaires aux ateliers de maintenance, les autorités organisatrices pourront en récupérer la propriété. Pour ce qui est des gares, l'ouverture à la concurrence impose de séparer le gestionnaire des gares de l'opérateur historique de transport, SNCF Mobilités, afin de garantir aux entreprises ferroviaires un accès transparent et non discriminatoire aux gares de voyageurs. À cette fin, l'article 11 prévoit la transformation, au 1 janvier 2020, de Gares & Connexions en société anonyme à capitaux publics, filiale de l'établissement public « de tête » SNCF. Le capital social de Gares & Connexions pourra être ouvert à d'autres investisseurs, afin de contribuer au développement et à la modernisation des gares, l'État devant, en tout état de cause, demeurer l'actionnaire majoritaire. L'État conclura avec Gares & Connexions un contrat pluriannuel fixant des objectifs de gestion des gares, notamment en matière de trajectoire financière, de qualité de service et d'aménagement du territoire. Afin d'assurer l'indépendance des dirigeants de Gares & Connexions à l'égard des entreprises ferroviaires, plusieurs garanties sont prévues, sur le modèle de ce qui existe actuellement pour SNCF Réseau. Enfin, pour faciliter l'information aux voyageurs et la vente des billets dans le contexte de l'apparition de nouveaux opérateurs, l'État pourra imposer aux entreprises ferroviaires de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente des billets. Pour conclure, je veux me réjouir que nous puissions, ici, au Sénat, avoir un débat sur un sujet aussi important, qui a des impacts, on l'a vu, sur les usagers, comme sur les territoires. Le texte que nous examinons aujourd'hui a été préparé très en amont, après de nombreuses consultations. Il constitue un dispositif équilibré, dont nombre de mesures sont partagées par plusieurs acteurs du secteur. Mes chers collègues, comme le disait Gérard Cornu en commission, saisissons-nous de ce dossier relatif à l'aménagement du territoire et à la desserte de l'ensemble du territoire par les transports ! Je vous invite donc à soutenir cette proposition de loi.

Face aux transformations politiques, économiques et sociales qui bouleversent notre société, nos concitoyens, nos territoires ont besoin de mobilité.

Ces mobilités- professionnelle, culturelle ou sociale -dont notre société a tant besoin ont un préalable : la mobilité physique. Force est de constater qu'aujourd'hui les Français ne sont pas égaux face à la mobilité. L'absence de solutions de mobilité est encore trop souvent un frein pour l'accès à l'éducation ou à l'emploi. Elle alimente un sentiment d'assignation à résidence chez certains de nos concitoyens et d'abandon dans de trop nombreux territoires. Je ne peux m'y résoudre. Peut-on accepter que, dans notre pays, une personne sur quatre ait refusé un emploi ou une offre de formation en raison de difficultés de déplacement ? L'objectif du Président de la République et du Gouvernement est d'accompagner tous nos territoires, de répondre aux préoccupations premières de nos concitoyens et aux besoins des entreprises : les transports du quotidien, la lutte contre la congestion des grandes agglomérations, l'accès à l'emploi et aux services dans les territoires, l'optimisation de nos systèmes logistiques. Dès lors, mon rôle, en tant que ministre des transports, ne se réduit pas à proposer une évolution, ici, du train, là, de la route ou bien des voies fluviales. Mon ambition consiste à redonner à nos politiques de mobilité un objectif très simple : répondre aux besoins de mobilité des Français. ces besoins, quels sont-ils ? Ce sont ceux qui sont exprimés par nos concitoyens, à Aurillac, à Prades, en passant par Strasbourg, lors des Assises nationales de la mobilité.

Nos concitoyens nous le disent : « Nous voulons des transports quotidiens efficaces. » Pour répondre à ce besoin vital, le système ferroviaire a toute sa place. Il joue, depuis bientôt deux siècles, un rôle central dans les déplacements de nos concitoyens, dans l'attractivité économique de notre pays et dans l'aménagement de nos territoires, dont il a largement contribué à redessiner la géographie. Parce que je suis convaincue que ce rôle doit rester au coeur de notre politique de mobilité, doit perdurer en se renouvelant, j'ai souhaité présenter une stratégie d'ensemble de refonte de notre système ferroviaire. En effet, alors que le système ferroviaire est, en quelque sorte, un ADN commun à tous les Français, force est de constater qu'il est à bout de souffle. Vous le savez, depuis une trentaine d'années, priorité a été donnée à la grande vitesse, incontestable succès technique et commercial, les statistiques de trafic pour 2017 le prouvent encore. Si la fonction d'aménagement du territoire de ces lignes à grande vitesse ne doit pas être minimisée, il subsiste pour autant de nombreux besoins insuffisamment satisfaits. Ces derniers étaient d'ailleurs au coeur de nos échanges cet après-midi. Par ailleurs, le transport ferroviaire de marchandises est en crise, avec des trafics inférieurs de 40 % à ceux du début des années 2000. C'est une situation dont toute une économie pâtit et à laquelle il faut une meilleure réponse. Enfin, le déséquilibre économique et financier du système non seulement pèse sur les finances publiques, mais menace également l'avenir du système ferroviaire ; je pense en particulier à la question de la dette. Vous le reconnaîtrez comme moi, tout ne marche donc pas au mieux dans notre système ferroviaire actuel. Comment produire des mobilités vertueuses et efficaces quand les vitesses de circulation sont actuellement ralenties sur plus de 20 % du réseau, soit deux fois plus qu'il y a dix ans ? Et que penser alors de la dette que je viens d'évoquer, qui se creuse de 3 milliards d'euros chaque année, pour atteindre 50 milliards d'euros aujourd'hui ? Faire comme en Allemagne ! Aussi, le Président de la République et le Gouvernement portent un projet ambitieux pour notre système ferroviaire français cette réforme globale doit construire les bases durables d'un meilleur service public ferroviaire ; en d'autres termes, l'objectif est d'avoir un meilleur service public, au meilleur coût, pour les voyageurs et les contribuables. Concrètement, cela veut dire : pour les voyageurs, des trains plus ponctuels, plus de trains là où il y en a besoin, avec plus de services, et en toute sécurité pour la SNCF, un modèle économique enfin équilibré, une entreprise publique plus forte, avec tous les atouts pour faire face à la concurrence ; pour les cheminots, une vision claire de l'avenir, avec des métiers attractifs et une reconnaissance de leur rôle pour les contribuables, la garantie que chaque euro pour le service public ferroviaire est dépensé efficacement. Afin d'y parvenir, nous devons mener une réforme cohérente, articulée sur deux engagements forts de l'État. Le premier, celui d'investir plus qu'il ne l'a jamais fait pour le ferroviaire : 36 milliards d'euros dans les dix prochaines années pour les infrastructures, soit 50 % de plus que sur la dernière décennie. Le second, celui de donner un nouveau cadre au ferroviaire, pour une ouverture à la concurrence réussie et stimulante pour la SNCF. En cela, la question de la transformation en société nationale à capitaux publics ne doit pas être un tabou. Je m'engage de nouveau solennellement sur ce sujet devant la Haute Assemblée : la SNCF est une entreprise publique, et elle le restera. Dans le même temps, la SNCF doit conduire sa réforme, au travers d'un nouveau projet d'entreprise, pour mieux répondre aux attentes de ses clients voyageurs et fret, en proposant un cadre social motivant pour les cheminots. Et c'est bien parce qu'elle doit avoir toute sa part dans notre nouvelle politique de mobilité qu'il est nécessaire de refonder la SNCF sur des bases modernes, agiles, unifiées, afin de préparer l'entreprise publique à relever ces nouveaux défis. Je veux dès maintenant le préciser : accompagner la SNCF dans le XXIsiècle, c'est également pour moi la conforter dans son rôle fondateur, au service de l'aménagement durable des territoires. Vous l'aurez compris, il n'est donc pas question de supprimer, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, les lignes de maillage et d'intérêt local, improprement appelées « petites lignes ». Il s'agira, au contraire, de faire en sorte que ces lignes puissent retrouver leur attrait et soient en mesure de répondre aux besoins. De même, le modèle d'un TGV assurant une desserte des villes moyennes au-delà des lignes à grande vitesse doit être conforté par la réforme. Là encore, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux être claire : personne ne remet en cause ce modèle. Nous pourrons débattre de la méthode retenue dans la proposition de loi et des alternatives possibles. de cette réforme, la question de l'ouverture à la concurrence est naturellement essentielle. La proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner la soulève avec une juste acuité. Je Je voudrais saluer la qualité des travaux engagés de longue date par votre Haute Assemblée sur cette question, par votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, son président, son rapporteur et votre ancien collègue Louis Nègre. Effectivement, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui rejoint, sur certains points, les thèmes que le Gouvernement entend traiter dans le projet de loi pour un « nouveau pacte ferroviaire Pour autant, vous le savez, la concurrence n'est qu'un des éléments du projet présenté le 26 février dernier par le Premier ministre. Parce qu'elle repose sur une volonté forte, celle de répondre aux besoins de nos concitoyens et de nos entreprises, parce qu'elle ne refuse pas de prendre à bras-le-corps les difficultés que rencontre notre système ferroviaire, parce qu'elle entend répondre aux inquiétudes exprimées par les cheminots, vous l'aurez compris, l'ambition du Gouvernement de remettre sur pied notre système ferroviaire ne se réduit pas à l'ouverture à la concurrence. Le pacte ferroviaire porté par le Gouvernement se place dans une vision plus large des mobilités au service du pays. Il s'inspire de la richesse des échanges des Assises nationales de la mobilité et de la rigueur des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Il s'inscrit dans une démarche globale permettant, trente-six ans après la loi d'orientation sur les transports intérieurs, de redéfinir l'ensemble des outils de notre politique de transport. Je pense, par exemple, à la constitution d'autorités organisatrices dans les territoires qui en sont actuellement dépourvus, à la création de leviers pour encourager toutes les initiatives pertinentes et efficaces permettant de proposer des solutions de mobilité ou à la programmation sincère de nos investissements en termes d'infrastructures. termes d'infrastructures. J'en viens à la méthode choisie par le Gouvernement. Elle a, je le sais, suscité des interrogations auxquelles l'inscription de cette proposition de loi me donne opportunément l'occasion de répondre. Le projet de loi que je porte n'entame pas le temps du dialogue social, bien au contraire. J'ai engagé un processus de concertation et de négociation avec l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des organisations syndicales, bien sûr, mais également des représentants des usagers, des entreprises ou encore des collectivités concernées. Cette réforme suscite, vous le savez, de légitimes interrogations chez les cheminots. C'est dans la concertation et par le dialogue que nous pourrons y répondre. J'ai démarré cette concertation voilà quatre semaines. Nous avons déjà tenu plus de quarante réunions, près de soixante-dix sont d'ores et déjà prévues, et elles sont indispensables. Le projet de loi que je porte n'entame pas non plus le temps du débat parlementaire. Comme je m'y suis engagée, il sera enrichi des concertations en cours afin qu'elles puissent être débattues et votées au Parlement. À cet effet, chaque fois que nous aurons suffisamment avancé dans la concertation, nous introduirons, par voie d'amendement, les dispositions correspondantes à la place des ordonnances. Le Parlement ne sera pas privé d'un débat de fond, au fond ou plutôt à la hauteur des enjeux de cette réforme. La richesse des échanges que nous aurons ce soir, qui se poursuivront demain et dans les prochains jours sur le projet de loi que je vous présenterai, en portera témoignage. Alors que les discussions avec les organisations syndicales et patronales ne sont pas encore terminées- convaincue de votre attachement au dialogue social -, vous comprendrez que le Gouvernement ne puisse se prononcer aujourd'hui sur l'ensemble de cette proposition de loi. Cela étant, je ne doute pas que plusieurs dispositions de la présente proposition de loi viendront enrichir le texte que je porterai au cours de la navette.

un patrimoine vivant de l'engagement quotidien des femmes et des hommes qui y travaillent avec passion : les cheminots. Cet héritage commun, ce bien public, je souhaite non seulement le préserver, mais également le conforter, pour répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens et des territoires.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quelques jours après la première grande manifestation à Paris pour la défense du service public, nous engageons, avec l'examen de cette proposition de loi, la première étape parlementaire de la réforme ferroviaire. Je le dis d'emblée, les sénatrices et sénateurs de mon groupe soutiennent tous les agents du service public, qui oeuvrent chaque jour, et même chaque nuit, pour que notre droit à la mobilité soit garanti. Ces agents exigent, avec dignité, le respect du dialogue social et la préservation de leur outil de travail. Nous serons donc à leurs côtés dans toutes les actions collectives qu'ils décideront de mener pour s'opposer à la casse du service public ferroviaire. Venons-en à cette proposition de loi. Le Gouvernement, qui fait peu de cas des institutions démocratiques, dont le Parlement, a fait le choix de passer son « nouveau pacte ferroviaire » par ordonnances et dans la précipitation. Pour répondre à cette provocation, la conférence des présidents du Sénat a fait le choix d'inscrire à notre ordre du jour, en urgence également, la présente proposition de loi, pour qu'elle devienne le support législatif de ce nouveau pacte ferroviaire. ferroviaire. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que le ferroviaire est un sujet trop structurant pour nos territoires pour le laisser à la seule discrétion du pouvoir exécutif. La représentation nationale doit pouvoir exercer ses prérogatives. Cette posture gouvernementale se double d'une certaine idée du dialogue social, cette méthode étant utilisée comme un moyen de faire pression sur les partenaires sociaux. Le chantage est le suivant : soit vous êtes raisonnables et l'on transforme progressivement les ordonnances en dispositions législatives ordinaires, soit vous vous obstinez, et tout vous échappera. Nous partageons donc pleinement la volonté du Sénat de signifier au Gouvernement notre refus de légiférer par ordonnances sur un tel sujet, notre refus de voir le dialogue social si malmené. Nous Nous exprimons aussi l'idée qu'il faut donner le temps nécessaire au travail législatif. Cependant, sur ce point, nous sommes un peu gênés : même si nous comprenons l'urgence d'une réponse rapide du Sénat, celle-ci conduit dans les faits à malmener les droits des parlementaires. La proposition de loi ayant été inscrite à l'ordre du jour voilà deux semaines, il est impensable de demander aux parlementaires, à ceux des petits groupes, un travail législatif rigoureux dans des délais si contraints. Ces délais contraints se conjuguent en outre avec un déficit d'information. Sur un tel sujet, il nous semble indispensable de disposer d'une étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État.

tout en ne partageant pas le message envoyé aux sénatrices et sénateurs appelés à adopter cette proposition de loi comme un élément de contestation, mais sans avoir à se prononcer sur son contenu. Or, sur le fond, nous nous trouvons face à une variation sur un même thème, celui du quatrième paquet ferroviaire, qui entérine l'ouverture à la concurrence des transports de voyageurs, lignes à grande vitesse comme trains régionaux. Les sénateurs du groupe CRCE sont radicalement opposés à cette démarche qui condamne le service public ferroviaire. il est illusoire de penser que l'on peut marier une politique d'aménagement du territoire avec la libéralisation du rail, qui conduit à des politiques de court terme, centrées sur la rentabilité de l'offre. Nous y opposons l'intérêt général, la réponse aux besoins exprimés en termes d'aménagement du territoire, de droit à la mobilité ou de transition environnementale. Nous considérons ainsi- c'est ce qui motive cette motion -que cette proposition de loi ne doit pas être le support de la réforme ferroviaire. En premier lieu, nous estimons que les directives européennes sont faites pour être révisées si elles ne répondent pas à leur postulat de départ, en l'occurrence une amélioration du service. Nous estimons ainsi que la France, forte de son expérience en matière d'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, laquelle s'est traduite par un recul du rail au profit de la route, une rétraction du réseau- et même son abandon parfois - ainsi que la fermeture de triages, devrait pouvoir demander la renégociation de l'ensemble des paquets ferroviaires. les expériences étrangères nous démontrent que cette voie n'est pas souhaitable pour les usagers. En effet, les tarifs explosent, comme on le voit en Grande-Bretagne, sans compter les aspects de sécurité ferroviaire, celle-ci étant bien plus difficile à obtenir avec la multiplication des opérateurs. la proposition de loi comporte des éléments particulièrement inquiétants, qui vont plus loin que les exigences du quatrième paquet ferroviaire. Tout d'abord, elle anticipe les dates d'ouverture à la concurrence des transports conventionnés. le droit européen est muet sur le régime de propriété des entreprises qui assument un service public. Il n'est aucunement exigé par le droit européen que Gares & Connexions change de statut. C'est une décision purement idéologique, partagée d'ailleurs par le Gouvernement, qui souhaite changer le statut de l'ensemble de l'entreprise publique. Pour notre part, nous sommes opposés à tout changement de statut. Nous considérons que la forme publique est la plus adaptée à l'exercice du service public. En l'occurrence, les gares sont des structures d'aménagement du territoire qui ne doivent appartenir qu'à la puissance publique, sous une forme garantissant cette pleine maîtrise publique.

SNCF. Nous nous trouvons, là aussi, face à une posture idéologique. Même le projet gouvernemental est plus souple, en retardant l'ouverture en Île-de-France du fait de la densité des réseaux. Nous pensons, pour notre part, que ces exceptions pourraient être invoquées pour l'ensemble des régions. Concernant les modalités d'ouverture à la concurrence, j'entends

c'est mieux que l'prévu par le Gouvernement, mais nous restons dubitatifs. Pouvez-vous réellement nous assurer que, malgré ce redécoupage, certaines lignes ne seront pas purement et simplement abandonnées ? De plus, quelles que soient les modalités choisies, c'est bien la cohérence globale de l'offre de transport qui perd du sens et de la pertinence. Avec un service qui sera à géométrie variable en fonction de la région habitée, des territoires entiers regarderont Cette ouverture à la concurrence sous toutes ses formes ouvre donc bien la voie à la balkanisation du service public ferroviaire et de la SNCF, une posture fortement accidentogène qui va perturber la cohérence du système ferroviaire. Concernant le statut des cheminots, l'attaque est moins frontale que celle du rapport Spinetta, mais elle est pernicieuse. Le transfert des salariés aux autres entreprises ferroviaires n'est pas encadré. Aucune obligation préalable n'incombe à la SNCF en matière de reclassement. Une sorte de portabilité des droits est mise en place, mais comment la garantir sur le long terme par des entreprises privées ? La possibilité de licencier un cheminot qui refuserait son transfert est incompatible avec le statut des cheminots, qui garantit la continuité du service public, et donc de l'emploi. Au final, il existe plusieurs points communs entre toutes ces propositions, projets de loi et rapports. Deux constantes peuvent être relevées : l'ouverture à la concurrence et l'idée qu'il faut en finir avec toute notion publique dans les transports ferroviaires. Nous nous inscrivons en faux contre cette vision qui se place d'un strict point de vue organisationnel, structurel et financier. Nous considérons que, pour faire une réforme efficace, il convient d'abord de prendre en compte les besoins. Or les usagers n'ont pas besoin d'avoir le choix, ils ont besoin d'avoir des trains qui fonctionnent, qui soient ponctuels, en nombre suffisant et en tous points du territoire. Pour cela, il faut s'atteler aux véritables maux qui affectent le service public ferroviaire : le sous-financement chronique des infrastructures, la charge de la dette, qui obère les capacités d'investissement, l'abandon de certaines dessertes ou de certaines activités sur des critères comptables, ou encore l'avantage concurrentiel de la route. Aujourd'hui, il nous semble important de soutenir le service public ferroviaire, en trouvant de nouvelles sources de financement, en retrouvant une politique de massification et de développement de l'offre et en supprimant les avantages pour la route, notamment par le retour d'une écotaxe poids lourds. Il nous semble nécessaire de s'intéresser aux politiques d'aménagement pour éviter de créer toujours de nouveaux besoins de mobilité par l'étalement urbain et de réfléchir à de nouvelles complémentarités entre les différents modes de transport. Il convient de renforcer les péréquations au lieu d'organiser la balkanisation des opérateurs et des territoires. La régionalisation, renforcée par ce projet de loi, est une impasse, y compris pour les régions elles-mêmes,

la transition environnementale et de se doter des outils permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour respecter les engagements de l'accord de Paris. Autant de problématiques absentes de cette proposition de loi ! Voilà les raisons qui nous ont conduits à déposer cette motion.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, je prends la parole contre cette motion, car il me paraît incompréhensible de fustiger la volonté du Gouvernement de légiférer par ordonnances sur la réforme de notre système ferroviaire,

Ce refus de débat est préjudiciable à l'expression démocratique et à la Haute Assemblée, qui utilise pleinement le pouvoir d'initiative donné aux parlementaires par la réforme constitutionnelle de 2008, laquelle a vraiment renforcé le pouvoir du Parlement. La proposition de loi que nous examinons a été préparée par le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey, et notre ancien collègue, Louis Nègre, grand spécialiste des questions relatives aux transports, au cours de l'année 2017. Elle a pour objet de définir un cadre juridique adapté à la réforme ferroviaire, sans en anticiper les échéances. À l'origine, cette initiative visait à permettre aux parties prenantes de se préparer en amont, alors que l'insuffisante préparation de la libéralisation du fret ferroviaire a eu, nous le savons tous, des conséquences très négatives, surtout pour l'opérateur historique. Pour préparer ce texte, les auteurs ont recueilli, lors de plusieurs dizaines d'heures d'auditions, les positions des différents acteurs concernés : les usagers, les syndicats, les régions, l'ARAFER, l'Autorité de la concurrence, le groupe public ferroviaire, les nouveaux entrants, les ministères concernés. Ils ont aussi entendu des universitaires et ont ensuite procédé à une consultation par voie écrite. Cette proposition de loi a été déposée le 6 septembre 2017. À la demande du président du Sénat, elle a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État, rendu le 22 février 2018 et publié, ce qui est rare. Cette procédure a permis d'identifier les améliorations possibles du texte sur le plan juridique. Le travail en commission, avec l'adoption d'amendements inspirés de l'avis du Conseil d'État, nous a permis d'aboutir à un texte juridiquement solide. Il nous paraît donc important que nous puissions examiner cette proposition de loi, afin d'avoir un vrai débat parlementaire, chose que le projet de loi d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances, je le répète, ne nous permettra pas. Mes chers collègues, par de nombreux aspects, notre système ferroviaire a été une réussite un vaste réseau, une grande vitesse très développée, un transport régional et local dense. Et nous savons combien le transport ferroviaire peut être facteur de compétitivité, d'attractivité pour nos territoires et gage de mobilité pour tous Malheureusement, à la veille de l'ouverture à la concurrence, les performances de notre système ferroviaire apparaissent clairement insuffisantes et nécessitent modernisation et adaptation. adaptation. La qualité de service s'est dégradée au fil des années et plusieurs accidents majeurs ont également terni l'image du groupe public ferroviaire en matière de sécurité. Le réseau demeure vieillissant, malgré les travaux de régénération. Après vingt ans de réformes successives, notre système ferroviaire ne semble toujours pas prêt pour la concurrence. Pourtant, il y a urgence. Le quatrième paquet ferroviaire, adopté en deux temps dans le courant de l'année 2016, généralise le droit d'accès au réseau, jusqu'à présent réservé aux services internationaux de transport de voyageurs et aux dessertes intérieures effectuées dans le cadre de ces services, à l'ensemble des services de transport de voyageurs à partir du 1 janvier 2019, pour une application effective à partir du 14 décembre 2020, soit au début de l'horaire de service 2021. De plus, ce texte européen enjoint les États membres à en assurer la transposition au plus tard le 25 décembre 2018. Il est donc urgent de fixer le cadre juridique de l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires, conventionnés ou non, non seulement pour respecter les échéances européennes, mais aussi pour permettre aux différentes parties prenantes, y compris l'opérateur historique, de s'y préparer dans des conditions convenables, tant pour ses personnels que pour les usagers. Nous ne pouvons plus faire la « politique de l'autruche » en nous focalisant sur des dérogations ou en feignant de ne pas voir que, si la concurrence progresse partout en Europe sur le trafic intérieur des États membres, la France ne pourra rester isolée, isolée, lorsque la SNCF opère sur les marchés étrangers en étant compétitive ! Nous le savons bien, cette ouverture à la concurrence sera sans doute limitée et progressive, mais la prudence et la lucidité obligent tous les opérateurs à s'y préparer. La concurrence de sociétés privées sur le marché ferroviaire ouvert aura des conséquences pour la SNCF, mais il n'y a pas de raison pour que la SNCF ne profite pas, à son tour, de l'ouverture, en assurant des dessertes intérieures dans d'autres pays. Par ailleurs, si le réseau à grande vitesse est d'ores et déjà ouvert à la concurrence sur les lignes internationales depuis plusieurs années, qu'il s'agisse de Paris-Bruxelles ou de Paris-Londres, aucun concurrent ne s'est manifesté ... L'ouverture du marché peut donc être source de gains si l'entreprise SNCF On le voit, tous les pays qui ont mené des ouvertures à la concurrence réussies ont, en parallèle, mis en place les conditions d'un équilibre économique global du système ferroviaire et ont renforcé sa gouvernance. La France n'a toujours pas effectué cette nécessaire « remise à plat », avec une dette ferroviaire qui continue d'augmenter, un effort de modernisation qui reste insuffisant et des services qui pourraient être renforcés dans certaines zones. Cette nouvelle réforme du système ferroviaire français semble donc plus que nécessaire. L'ouverture à la concurrence, que nous appelons de nos voeux, permettra, nous en sommes convaincus, de renforcer la compétitivité de l'opérateur historique et sera également bénéfique aux usagers du transport ferroviaire comme aux contribuables français. Pour toutes ces raisons, nous désapprouvons cette motion de procédure, qui marque le refus de poursuivre le débat sur un sujet essentiel pour notre pays.

nous estimons indispensable d'avoir un débat parlementaire sur la mise en oeuvre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, une réforme majeure ayant des impacts sur les personnels, les usagers et les territoires.

Au-delà de ce sujet, d'autres questions importantes doivent être traitées. Les conditions de transfert des personnels en cas de changement d'opérateur- nous examinerons ce propos un amendement présenté par notre collègue Gérard Cornu à l'article 8 -, la gestion des gares, les conditions de transmission des informations nécessaires aux autorités organisatrices, la propriété des matériels roulants et des ateliers de maintenance, la vente des billets ainsi que l'information aux voyageurs

l'avis du Gouvernement ? Comme je l'ai indiqué, le Gouvernement propose une réforme ambitieuse. Le projet de loi, qui a été présenté en conseil des ministres le 14 mars dernier, fait actuellement l'objet de concertations. Cette réforme globale et cohérente repose sur quatre axes : améliorer le service public, avec un programme d'investissements massifs pour remettre à niveau un réseau qui souffre de décennies de sous-investissement préparer une ouverture progressive à la concurrence des TER et des TGV ; mettre en place un cadre social protecteur et équitable, pour tenir compte

équilibré. Le Gouvernement aborde ce débat avec une volonté d'écoute et d'échanges, mais il ne pourra pas se prononcer sur l'ensemble de la proposition de loi. Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur la motion présentée.

Le scrutin est ouvert.

la SNCF, ce monument des services publics qui a tant fait pour notre République, notamment pour son unité, grâce à son réseau en étoile. Merci, donc, à MM. Maurey et Nègre, que je salue, d'avoir su préparer une réflexion qui a de l'intérêt et qui anticipe efficacement l'échéance du 25 décembre 2018. de ce texte est de nous permettre de débattre du ferroviaire. Ce débat a été confisqué par le Premier ministre, le 26 février, lorsqu'il a annoncé que le Gouvernement recourrait aux ordonnances, alors même que, contrairement à la réforme du code du travail, le Président de la République n'en avait pas parlé lors de sa campagne présidentielle. Je m'interroge quant à ce contournement délibéré des chambres ... Conséquence directe de cela, madame la ministre, vous nous avez conduits à agir en comme vient de le dire Hervé Maurey, alors que cette proposition de loi était prête fin 2017 et que cette échéance de fin 2018 est connue depuis deux ans. Je note par ailleurs que la réforme de 2014 a été utile, appréciée, et même salutaire, et qu'elle n'a pas eu besoin d'ordonnances. Nous pourrions apporter les améliorations aujourd'hui nécessaires de cette même manière. Votre intention de départ était pourtant louable. Vous nous proposiez, en juillet, une belle et grande loi sur les mobilités, à la hauteur de la LOTI de 1982, consacrant la nouvelle logique de mobilités, plutôt que de transports, et proposant l'intermodalité, l'interconnexion et la conjugaison des modes afin que nos concitoyens puissent relier efficacement et écologiquement un point A à un point B. Vous nous aviez d'ailleurs mis l'eau à la bouche avec les intéressantes Assises nationales de la mobilité. de la mobilité. La SNCF et le ferroviaire ont besoin d'un véritable débat démocratique et non pas de concertations en marge d'ordonnances. Vous vous attaquez là à une institution totémique, au patrimoine commun des Français. Pis, le Premier ministre a voué la SNCF et les cheminots aux gémonies, mettant le mythique statut en pâture, faisant croire qu'il serait le problème. Le problème, nous le savons, il réside aujourd'hui pour l'essentiel dans cette dette considérable, cette dette qui n'est pas celle des cheminots, mais bien davantage celle des différents gouvernements, qui, depuis des décennies, envoient des injonctions contradictoires à la SNCF, lui intimant plus d'économies et, en même temps, plus d'investissements pour les LGV, et ce au détriment de l'entretien des réseaux. Le problème, il est aussi dans le financement des infrastructures et de la tarification

est un héritage et un patrimoine considérables ; nous ne pouvons l'évaluer à l'aune des seules annualités budgétaires. Nous devons prendre en compte la transition écologique, la pollution, les congestions automobiles et l'ensemble des services rendus. aussi l'aménagement du territoire, puisque c'est aussi et presque surtout de cela qu'il s'agit. Si les régions sont les chefs de file incontestés en matière de transport depuis la loi NOTRe, c'est bien par elles que passera le développement des offres de mobilités de demain. Votre volonté de leur confier la gestion des lignes de catégorie 7 à 9 sans imaginer, pour le moment, les moyens financiers pour les faire vivre revient de fait à les condamner. Nous ne pouvons pas nous résoudre à abandonner la ruralité en sacrifiant les gares après les bureaux de poste J'en viens à la proposition de loi sur laquelle nous allons être amenés à nous prononcer. Elle a le mérite, je le répète, d'ouvrir la discussion sur le sujet du ferroviaire, mais elle a le défaut de nous propulser dans une situation d'urgence pire encore que celle des ordonnances. Nous avons eu à peine quinze jours

Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si nous sommes pour ou contre l'ouverture à la concurrence. Le quatrième paquet ferroviaire l'a tranchée.

Nous préférons dynamiser plutôt que dynamiter ! Je ne tiendrai pas un discours manichéen sur le sujet de l'ouverture à la concurrence. elle a pu bien fonctionner dans certains pays et être catastrophique dans d'autres, l'un des pires exemples étant la libéralisation du fret ferroviaire dans notre pays en 2006, mal préparée, mal évaluée, mal anticipée. Résultat : un effondrement du volume de transport et une explosion du nombre de camions sur nos routes, déjà trop nombreux à l'époque. Pas de dogme,

de nos concitoyens. Autre constat qui montre que tout n'est pas noir : depuis 2004 et la régionalisation, le nombre de passagers des TER a augmenté de 44 % et l'offre a été décuplée, et ce malgré un dialogue parfois difficile entre nos collègues élus régionaux, la SNCF et ses différentes composantes. Une fois que la loi sera votée, il faudra du temps aux acteurs, aux autorités organisatrices et aux opérateurs pour bien préparer l'ouverture raisonnée à la concurrence. C'est pourquoi il nous semble primordial de garder 2023 comme date limite d'ouverture à la concurrence pour les régions tant les situations sont diverses.

nous serons nuancés et prudents devant votre proposition reprenant le principe dominant des franchises, philosophiquement intéressant, mais dans les faits difficile à mettre en oeuvre, aux niveaux tant de la répartition des lots que des continuités de service entre eux. Il pourrait également impacter fortement l'opérateur actuel. Le libre accès, pour autant, nécessite de très fortes régulations, qui restent encore à imaginer, pour éviter l'écrémage. Il y aura certainement des candidats pour reprendre le Paris-Nancy, qui voudra de son prolongement vers Mirecourt, voulu par les élus locaux et le président Poncelet ? Concernant le personnel, cette proposition de loi a été rédigée avant que le Premier ministre n'annonce la fin du statut pour les nouveaux recrutements. Il y aura à dire ! Je note que, s'agissant des mouvements entre opérateurs, il est proposé ici de garantir les conditions d'origine au-delà du premier transfert, là où le rapport Spinetta ne parle que du premier transfert. En revanche, nous nous inquiétons du durcissement de la législation actuelle, qui est inscrite à l'article 8. Si le mythique statut prémunit les cheminots contre le licenciement économique, ils peuvent d'ores et déjà être licenciés en cas de refus de mobilité, mais seulement au bout du troisième refus. Nous ne pouvons donc accepter une disposition visant à mettre fin au contrat de travail dès le premier refus. Vous proposez également de rendre publiques les données de la SNCF, y compris celles qui seraient couvertes par le secret industriel ou commercial. Nous présenterons un amendement dont l'adoption permettrait, je pense, de mieux garantir le risque de fuites de données essentielles vers les concurrents de notre opérateur actuel. Il en va de même concernant le matériel roulant ou les ateliers de maintenance. Il conviendra de veiller à un meilleur équilibre entre deux risques : celui qui verrait la SNCF devoir gérer seule les parties les moins intéressantes et celui qui verrait les nouvelles autorités organisatrices hériter d'une charge trop lourde. Nous avons besoin d'approfondir la question. et pas des moindres : les gares. Nous nous inquiétons de la volonté de transformation de l'entité Gares & Connexions en société anonyme. Nous plaidons résolument pour le maintien de la maîtrise publique des gares. Elles font partie du patrimoine national.

mais nous le voyons comme un hors-d'oeuvre, un galop d'essai avant d'aborder le contenu des futures ordonnances et des textes importants à venir en matière de mobilité. c'est bien ainsi qu'il faut aborder la question : sortir de la logique des transports pour entrer dans celle des mobilités du XXI siècle. Sur ces sujets, nous nous positionnerons selon trois axes de progrès. D'abord, il y a l'aménagement du territoire et la poursuite de la décentralisation. Ces réformes doivent permettre plus d'égalité entre les hommes et entre les territoires, car il n'y a pas de petits territoires : il y a la République française ! Ensuite, il convient de respecter les cheminots et les travailleurs des transports. Alors que certains rêvent de précarisation et de dumping social, nous pensons qu'il doit y avoir une véritable continuité dans la protection des travailleurs des transports, qu'ils soient dans un train, un tram, un bus. Je vous pose la question, chers collègues pourquoi ne pas imaginer une convention collective des transports terrestres ? Enfin, nous nous battrons pour conserver une maîtrise publique des services publics : pas question de brader au plus offrant notre patrimoine commun ! Alors, je vous le répète, il nous faut dynamiser, sans dynamiter ! La parole

ans, un peu plus même, le 1 septembre 1937, la presse française annonçait fièrement la création prochaine de la Société nationale des chemins de fer français, Créée par un décret-loi du Front populaire et effectivement mise en place en janvier 1938, cette société fusionnait les activités et le personnel de l'État, les grandes compagnies ferroviaires privées et les réseaux d'Alsace-Lorraine administrés par l'État. L'aventure ferroviaire tricolore entrait dans une nouvelle ère de son histoire. « La convention assurer une heureuse conciliation entre l'autorité de l'État et le maintien nécessaire des souples méthodes de gestion [ ...] d'un grand service industriel et commercial », expliquait Camille Chautemps, chef du gouvernement, gouvernement, à. Aujourd'hui, la convention semble définitivement remise en question. Le groupe est durablement endetté, la qualité de service fortement discutée et le grand public s'exaspère des grèves et de retards à répétition. D'abord, le groupe ferroviaire est aujourd'hui dans une situation financière catastrophique. Si la SNCF a présenté d'excellents résultats en 2017, avec une hausse de 4,2 % de son chiffre d'affaires, à 33,5 milliards d'euros, et un bénéfice net de 1,33 1,33 milliard d'euros, la dette est abyssale : 46,6 milliards d'euros pour SNCF Réseau et 7,9 milliards d'euros pour SNCF Mobilités. Pour beaucoup d'analystes, cette dette constituerait même un risque pour le contribuable. Madame la ministre, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas ignorer cet état Ensuite, la situation de ce groupe ferroviaire n'est plus tenable. Le rapport Spinetta, remis au Gouvernement mi-février, tire la sonnette d'alarme sur des réformes nécessaires fin du statut de cheminot et de ses avantages- garantie à vie de l'emploi, retraite anticipée, facilités de circulation, etc.

Surtout, la SNCF devra affronter demain l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs. Inutile de rappeler ce qu'un manque de préparation à l'ouverture à la concurrence signifierait pour ce secteur et pour la qualité du service, cela a déjà été fait lors d'un récent débat sur le secteur du fret ferroviaire. Nous sommes prévenus ! Le calendrier politique fait que l'examen de cette proposition de loi intervient quelques semaines avant le projet du Gouvernement. Devant l'urgence de la situation, il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités pour débloquer la situation et envisager l'avenir du rail français. Pour s'adapter et ne pas disparaître, la SNCF devra irrémédiablement changer. Alors, madame la ministre, mes chers collègues, pour paraphraser l'un des anciens présidents de la SNCF, Louis Armand, où en est le chemin de fer français ? Ce débat doit être l'occasion de poser de nouveaux jalons en prévision du projet de loi du Gouvernement. La proposition de loi nous semble intéressante, perfectible. Il nous paraît ainsi nécessaire de prendre en compte le besoin de maintenir les petites lignes au nom de la vitalité de nos territoires. En commission, sur proposition du rapporteur, notre collègue Jean-François Longeot, et avec un large soutien politique, nous avons introduit un nouveau mécanisme liant des contrats de lignes de TGV et des petites lignes. À l'avenir, cela doit être la norme. Oui à l'ouverture à la concurrence de nos lignes ! Oui, en même temps, à la continuité de nos politiques d'aménagement du territoire ! Notre groupe, vous le verrez, a d'ailleurs proposé un certain nombre d'amendements pour compléter cette proposition de loi. Ces amendements s'inscrivent dans une triple approche approche : protéger les territoires en introduisant dans la loi les dérogations autorisées par le règlement européen et en sollicitant l'avis de la Conférence nationale des territoires sur cette ouverture à la concurrence concurrence ; assurer une transition transparente et respectueuse de tous en privilégiant des politiques d'- le rapporteur en a parlé -et en programmant des points d'étape avec les représentants locaux ; enfin, saisir l'opportunité de réformer le régime ferroviaire en ne forçant pas les nouveaux entrants à reproduire les mécanismes aujourd'hui défaillants. sont, loin des caricatures, les trois piliers sur lesquels fonder la réforme du secteur ferroviaire.

à la veille de l'examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, nous nous réunissons aujourd'hui pour débattre de l'ouverture à la concurrence du deuxième plus grand réseau ferré d'Europe, après celui de l'Allemagne. Le Gouvernement propose de recourir aux ordonnances pour transposer le quatrième paquet ferroviaire et réformer la SNCF. La présente proposition de loi intervient donc à point nommé, car elle vient illustrer les vertus du bicamérisme, que le groupe du RDSE ne cessera de défendre, la qualité du travail sénatorial et la nécessité de garantir en toutes circonstances les pouvoirs du Parlement. Une réforme aussi majeure que celle du transport ferroviaire mérite cette discussion de fond, qui intéresse nos concitoyens non seulement en tant qu'usagers, mais aussi en tant que contribuables. Nous saluons ainsi l'initiative conjointe de notre collègue Hervé Maurey et de Louis Nègre, ancien sénateur.

D'autre part, la SNCF est confrontée à une dette importante et croissante- elle accumule 2 milliards d'euros par an de déficit -ainsi qu'à une stagnation de la part modale du ferroviaire depuis 2010. Nous préparons l'ouverture à la concurrence dans un contexte particulier : l'État stratège est totalement absent depuis plus de trente ans en ce qui concerne l'aménagement du territoire, que ce soit en matière de choix de dessertes ou de financement des infrastructures. Les inquiétudes des agents, des usagers, des territoires et des parlementaires que nous sommes sont donc pleinement justifiées. Des directives sont données, mais la feuille de route n'est pas toujours lisible.

Avec 13 milliards d'euros de dépenses publiques allouées chaque année au ferroviaire, nos collectivités territoriales et nos concitoyens sont en droit d'exiger un service complet et de qualité. Or le taux de retard demeure élevé par rapport aux autres pays européens. Certes, la SNCF n'a pas vocation à être bénéficiaire, puisqu'elle remplit une mission de service public vitale pour l'accès de tous aux transports, la réduction des gaz à effet de serre et le maillage territorial. J'y suis particulièrement sensible, comme tous les membres de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Toutefois, j'ai la conviction qu'un tel service peut aller de pair avec une gouvernance efficace et des finances assainies. L'achèvement de l'ouverture à la concurrence constitue l'occasion pour la France d'apporter les améliorations qui s'imposent à la gouvernance de notre système ferroviaire. Le législateur déterminera les modalités de cette libéralisation, mais nous pensons que ce débat aurait dû avoir lieu avant 2018, dernière année avant l'échéance fixée par le droit européen. En l'état actuel, deux positions semblent se dessiner quant aux modalités de l'entrée des nouveaux opérateurs sur le marché des LGV d'un côté, l', permettant à toute entreprise d'accéder au réseau sans appel d'offres ; de l'autre, un système de franchises qui régulerait cet accès afin de ne pas remettre en cause la péréquation existant entre les lignes rentables et les lignes déficitaires, au détriment de l'aménagement du territoire. Les deux options comportent leurs avantages et leurs inconvénients. C'est la raison pour laquelle nos voisins européens ont procédé à une combinaison des deux. Le rapport Abraham de 2011 évoquait de multiples possibilités entre les deux extrêmes. la proposition de loi font le pari de la concurrence pour le marché pour certaines liaisons à côté des lignes en. Le Gouvernement semble préférer ce dernier, tout en envisageant d'imposer des obligations de service public, comme le propose le rapport Spinetta, qui évoque une taxe de péréquation afin d'éviter l'écrémage que les élus ruraux craignent à juste titre. Mes chers collègues, il est extrêmement difficile d'anticiper les effets de la mise en concurrence ou d'établir des comparaisons au niveau européen tant les marchés diffèrent, la part modale du ferroviaire en Allemagne ou en Italie restant, pour le moment, inférieure à celle de la France. Si la concurrence peut être bénéfique en matière de qualité de service, nous nous interrogeons sur ses effets à l'égard des prix et de la préservation des lignes peu rentables. Élu d'une zone géographique où le mot « enclavement » a du sens, je ne peux que saluer cette volonté de maintenir les lignes secondaires et d'inciter les entreprises à les desservir. La coordination de l'offre de transports sur l'ensemble de nos territoires doit également être assurée. L'usager doit rester au centre de l'organisation des dessertes sans pâtir de la multiplication des opérateurs. À cet égard, je salue la proposition de création par le texte d'un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets. Nombreux sont les points qui restent à trancher et qu'une proposition de loi ne peut avoir l'ambition de résoudre : avenir du statut du cheminot, du groupe ferroviaire intégré ; avenir des infrastructures et des financements, ou encore de la dette de SNCF Réseau. Cependant, l'aperçu de la réforme proposée par le projet de loi ne semble pas non plus régler cette question. La présente proposition de loi constitue un prélude à un débat éclairé au sein de la Haute Assemblée, alors que le champ d'habilitation proposé par le Gouvernement demeure à ce stade imprécis. Ainsi, nous ne disposons pas de tous les éléments, notamment du plus essentiel de tous : l'issue des concertations avec l'ensemble des parties prenantes. Or cette réforme historique ne peut faire l'économie d'un dialogue fondamental. Le groupe du RDSE, tout en reconnaissant la qualité de la proposition de loi, s'abstiendra toutefois sur ce texte. La parole est à M. Gérard Cornu, pour le groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe les Républicains se réjouit de l'inscription à l'ordre du jour de la Haute Assemblée de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire.

par le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey, et notre ancien collègue, Louis Nègre. Je les félicite pour la grande qualité de leur travail, qui s'inscrit dans une tradition sénatoriale

À l'origine, cette initiative visait à permettre aux parties prenantes de se préparer en amont, alors que l'insuffisante préparation de la libéralisation du fret ferroviaire a eu, nous le savons tous, des conséquences négatives. Elle va surtout nous permettre d'avoir un vrai débat au Sénat sur notre système ferroviaire, un débat que le projet de loi d'habilitation du Gouvernement n'autorisera pas. En dépit de réelles réussites et de profondes transformations opérées ces dernières années, la SNCF fait face à des difficultés structurelles importantes : infrastructures vieillissantes, exploitation complexe, qualité de service insatisfaisante ou modèle économique déséquilibré. Au-delà des moyens financiers nécessaires pour maintenir ce patrimoine ferroviaire, le moderniser, nous devons avoir une vision pour notre entreprise publique. Compte tenu de l'ouverture prochaine du marché du transport ferroviaire de voyageurs à la concurrence et face à l'attente légitime de nos concitoyens, la SNCF doit impérativement se réinventer. Elle doit continuer de remplir la mission de service public qui lui est confiée et, plus généralement, faciliter la mobilité de tous les Français. J'y insiste, de tous les Français

Dans le cadre de cette réforme, les efforts devront être partagés. En effet, l'État doit prendre sa part de responsabilité afin d'assurer la viabilité économique du système ferroviaire. Trop souvent, par le passé, l'État a fait supporter à la SNCF l'insuffisance des financements publics, ce qui a provoqué un endettement colossal de cette Cette reprise de la dette sera un point crucial lors de l'ouverture à la concurrence. Aussi, madame la ministre, nous aimerions vous entendre sur ce sujet très important. L'ouverture à la concurrence peut être l'occasion d'optimiser le système de transport ferroviaire de voyageurs en s'inspirant de la réussite d'une telle réforme dans d'autres pays européens. Cette proposition de loi est donc une véritable occasion à saisir pour le Gouvernement. Elle présente deux avantages : légiférer plus rapidement et permettre un véritable débat parlementaire.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Victor Hugo a un jour déclaré : « Je suis réconcilié avec le chemin de fer, c'est décidément très beau. S'il est une ambition que nous partageons tous dans cet hémicycle, c'est bien de parvenir à cette réconciliation et de pouvoir, collectivement, écrire l'avenir de notre chemin de fer. Car, oui, le chemin de fer est une partie intégrante de l'histoire de notre pays ! Il a apporté une contribution éclatante à l'aménagement de notre territoire national, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Notre imaginaire collectif y est à jamais associé grâce à Émile Zola, à Jean Renoir ou à cette image inoubliable de Jean Gabin dans, sans oublier Claude Monet et ses versions de la gare Saint-Lazare.

mes chers collègues, nous partageons sur ces travées le même constat : notre système ferroviaire est malade, encalminé, et il est essentiel qu'il se réinvente et se régénère pour être un acteur du formidable chantier des mobilités du quotidien qui s'ouvre devant nous. Madame la ministre, vous avez fait de la lutte contre « l'assignation à résidence » une priorité. Nous partageons tous, ici, cette volonté, qui doit être un marqueur fort de ce quinquennat. Ce combat est celui de tous les acteurs de la mobilité et, au premier rang d'entre eux, du service public ferroviaire, à la seule condition qu'il soit à la hauteur du rendez-vous. Tel est bien là l'objectif premier que poursuit le Gouvernement avec le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, présenté le 15 mars dernier. donne l'occasion de mettre un terme au débat qui agite une partie des élus de notre assemblée quant à la confiscation du débat parlementaire qui en serait la conséquence. N'ayons pas la mémoire courte, mes chers collègues. Rappelons que de grandes réformes sociales, porteuses de progrès, ont emprunté le même chemin. La sécurité sociale en 1945, ou bien encore le temps de travail, l'établissement de l'âge de la retraite à soixante ans, la cinquième semaine de congés payés en 1982 en sont quelques exemples patents, mais il y en a d'autres. Nous aurons un véritable débat, sans tabou aucun, sur l'avenir de notre service public ferroviaire, sans éluder aucune question, ce qui a été trop souvent le cas toutes ces dernières années. Le débat aura lieu, et je ne doute pas un seul instant que le Parlement saura faire entendre sa voix. Dans ce contexte, nous pouvons donc nous interroger légitimement sur l'opportunité de l'examen de cette proposition de loi articulée autour de l'ouverture à la concurrence et qui laisse de côté bien des sujets essentiels pour l'avenir de notre service public ferroviaire. L'inscription rapide de ce texte à notre agenda peut être sujette, dans le contexte du moment, à bien des interprétations, mais je préfère m'en tenir au fond et ne pas entrer dans telle ou telle polémique stérile. Sur le fond, soyons clairs, nous ne rejoignons pas forcément la position des auteurs de la proposition de loi, qui souhaitent accorder « des droits exclusifs aux entreprises ferroviaires pour l'exploitation des services de transport ferroviaire à grande vitesse, en contrepartie de la réalisation d'obligations de service public définies en fonction des besoins d'aménagement du territoire Comment imaginer qu'un cadre aussi contraignant garantisse un service de qualité aux usagers et un aménagement équilibré du territoire ferroviaire sans proposer des contreparties financières qui devraient être versées à un moment ou à un autre ? sa faisabilité nécessiterait une mise en oeuvre de moyens humains et financiers qu'il semble bien impossible de mobiliser. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder l'exemple britannique. Nous partageons la volonté de mise en oeuvre d'un modèle, d'un cercle vertueux, qui sera profitable aux usagers, aux entreprises ferroviaires, à l'État, aux collectivités territoriales et à l'aménagement du territoire. Le libre accès, ou, est une réponse qui peut paraître, de prime abord, déstabilisante, mais elle est surtout dynamisante. Chacun convient en effet de la nécessité d'instiller un aiguillon pour stimuler les exploitants et leur éviter de s'endormir sur leurs droits exclusifs. Le libre accès relève d'un espace d'initiative et de liberté commerciale. Encore convient-il de le mettre en oeuvre dans le cadre d'une refonte de la politique tarifaire des péages et d'un rôle conforté, voire accru, du régulateur qu'est l'ARAFER. effet, nous parlons ici non de dérégulation sauvage, mais de prévisibilité tarifaire encadrée, qui permettra notamment aux opérateurs d'être des acteurs clés de la révolution et d'irriguer tout ou partie du territoire national à l'instar d'autres pays et du succès remporté sur des lignes pourtant condamnées si rien n'était fait. Plus de trains qui roulent, plus de gares desservies, c'est à coup sûr renforcer l'offre des mobilités dans le pays, dans un cadre tarifaire supportable pour tous. Le cadre tarifaire est une constante dans notre histoire nationale. Je ne résiste donc pas au plaisir de partager avec vous, mes chers collègues, ces mots d'Alphonse Allais : « Les tarifs des chemins de fer sont aménagés d'une manière imbécile. On devrait faire payer des suppléments pour les retours ... puisque les gens sont forcés de revenir. » Au regard du formidable débat qui nous attend et de la concertation que vous avez initiée avec toutes les parties prenantes, madame la ministre, cette proposition de loi est comme ce voyageur sur le quai qui regarde partir le train qu'il vient de manquer. Nous avons en effet devant nous un défi immense. Le débat sur l'avenir du service public ferroviaire, nous l'aurons. Nous y aborderons tous les points : la transformation souhaitée de l'EPIC, la gouvernance de la SNCF, le calendrier souhaitable de l'ouverture à la concurrence, ses conséquences sur le matériel,

Au final, parce que l'avenir de notre service public ferroviaire ne se résume pas à la seule question de l'ouverture à la concurrence, le groupe La République En Marche votera contre cette proposition de loi. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour le groupe

De fait, notre système ferroviaire a toujours compté parmi les meilleurs au monde. Par son maillage extrêmement dense, il est un facteur essentiel d'égalité entre les citoyens et d'unité territoriale. Il assure tant la vitalité des territoires français que la cohésion du pays. Alors que la fracture territoriale et la transition écologique comptent parmi les défis majeurs du siècle, il est primordial de préserver notre réseau et notre excellence ferroviaires. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, dans la même veine que le projet d'ordonnances gouvernementales que nous examinerons demain, constitue un retour en arrière malvenu. En effet, il y a près de quatre-vingts ans, la SNCF a été créée pour pallier les difficultés d'investissements et d'organisation du secteur ferroviaire. En 1937, pour mettre un terme à la myriade inopérante de petites compagnies privées, le Front populaire a décidé de les unifier en une seule compagnie nationale. Cette décision historique a conféré à la puissance publique un rôle essentiel de stratège qui permettra à la SNCF non seulement d'atteindre l'excellence, notamment avec la création du TGV, mais aussi d'achever le maillage du territoire et d'assurer une nécessaire péréquation entre les lignes rentables économiquement et les lignes rentables socialement. Aujourd'hui, c'est tout cela que menace l'ouverture à la concurrence imposée par la délétère idéologie néolibérale de l'Union européenne. Non contente de répondre aux exigences de Bruxelles, cette proposition de loi fait du zèle. J'en veux pour preuve la privatisation des gares dont ce texte porte les germes, privatisation qui affaiblira, sans qu'il soit permis d'en douter, la densité du réseau. Plus largement, selon une logique libérale bien connue de privatisation des profits et de socialisation des pertes, c'est tout le réseau secondaire qui restera à la charge du contribuable et est, à terme, menacé de disparition progressive. Une telle perspective est plus qu'alarmante quand on examine les nombreuses enquêtes d'opinion en France, aux États-Unis ou en Autriche, qui établissent une corrélation irréfutable entre l'éloignement d'une gare et le vote en faveur de l'extrême droite ou des populistes. Supprimer une gare, supprimer une ligne, c'est renforcer ce sentiment d'abandon qui mine la concorde nationale. Ainsi, on s'achemine plus vers le catastrophique modèle britannique de privatisation totale du système ferroviaire- sur laquelle veut revenir une grande majorité de la population de Grande-Bretagne -que vers les modèles japonais ou allemand, souvent pris en exemple d'une ouverture à la concurrence réussie. À y regarder de plus près, il faut souligner que, dans les deux cas, la puissance publique a conservé un rôle essentiel de stratège. Au Japon, après un investissement public massif dans le réseau, la compagnie nationale a été divisée en six compagnies en six compagnies régionales. La dette a été répartie intelligemment entre l'État et les compagnies rentables. Le désengagement de l'État est tout à fait relatif, puisqu'il exerce toujours un strict contrôle sur les tarifs des billets et subventionne les compagnies déficitaires qui ont en charge les territoires les moins densément peuplés. Une réglementation claire et exigeante a été mise en place en cas de fermeture de ligne. De fait, la concurrence est limitée aux seules lignes extrêmement rentables de la mégalopole japonaise. En Allemagne, l'ouverture à la concurrence s'est accompagnée de la prise en charge par l'État des 35 milliards de dette de la Deutsche Bahn et de 50 milliards d'investissements supplémentaires pour la rénovation du réseau. La Deutsche Bahn est restée une compagnie publique assurant une mission de service public. On le voit, ces deux pays ont assumé la reprise de la dette ferroviaire et des investissements massifs dans leur réseau avant la mise en concurrence. Or ni cette proposition de loi ni le futur projet gouvernemental n'envisagent cela. Ils ne répondent donc pas aux deux problèmes structurels de la SNCF : sa dette colossale et la vétusté de son réseau, l'autre fruits de la stratégie du tout-TGV, lequel a trop longtemps mobilisé des financements massifs et obéré les besoins du réseau du quotidien. Pour remédier à ces problèmes, notre groupe, en prenant toute sa place dans le débat, vous proposera des solutions concrètes, telle la renationalisation des autoroutes ou la mise en oeuvre d'une écotaxe afin de dégager des ressources pérennes pour la SNCF. En effet, comme toujours, nous abordons ce débat à l'envers. À rebours d'un enjeu comptable, nous affirmons un enjeu de service public ; une mission de service public de proximité, assurée par des agents dévoués, qui ne sauraient être les épouvantails des difficultés de la SNCF et qui doivent, contrairement aux attaques pernicieuses que contient cette proposition de loi, être confortés dans leur statut. Loin d'être des privilèges, leurs acquis sociaux devraient être la norme pour toute travailleuse et tout travailleur de ce pays. En cette journée de célébration de l'héroïsme français, on rappellera opportunément que la convention collective des cheminots doit beaucoup à leur engagement fondamental dans la Résistance. dire que la réflexion sur l'avenir de la SNCF doit partir des besoins et non des moyens : du besoin de mobilité de tous nos territoires, nous l'avons dit, et du besoin impérieux de transition écologique. Si l'on excepte le matériel vétuste, le ferroviaire est de très loin le mode de transport le moins émetteur de gaz à effet de serre. Deux ans après la signature de l'accord de Paris, comment peut-on encore envisager de remplacer des trains par des cars ? Comment peut-on encore envisager de remplacer des trains de fret par des poids lourds sur nos routes, conséquence systématique de la libéralisation du rail ? Vous l'aurez compris, de notre point de vue, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes actuels du rail français. Pis, elle risquerait de les aggraver ! Sans surprise, le groupe CRCE ne la votera pas.

je tiens, en préambule, comme les orateurs qui m'ont précédée, à remercier MM. Hervé Maurey et Louis Nègre, qui, par cette proposition de loi, nous placent dans une démarche vertueuse d'anticipation de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire français. Une attitude frileuse, une attitude de blocage ou un manque d'anticipation pourraient nous faire manquer ce qui doit être une opportunité. Si nous attendons en rentrant la tête dans les épaules une ouverture subie comme une contrainte, nous regarderons passer le train, ce qui est un jeu de mots facile Au contraire, et puisque nombre d'entre nous n'ont guère envie de plaisanter sur le sujet, il faut que cette ouverture à la concurrence conduise à une amélioration du service pour les usagers et à une réduction des coûts. Il faut que ce changement soit une stimulation positive et saine, y compris pour l'opérateur historique. Voilà le fond de ce texte, et il ne peut faire que l'unanimité ! Cela étant, nos débats posent une question de forme sur laquelle je souhaite revenir pour clarifier la position du groupe Union Centriste. Centriste. Le Gouvernement, qui invoque des arguments de calendrier, propose de légiférer par ordonnances. Or nous venons de perdre des mois précieux qui auraient dû être destinés à un travail de fond collectif sur ce sujet capital. de loi d'Hervé Maurey et de Louis Nègre a en effet été déposée au mois de septembre. Il s'agit d'un texte abouti, qui a d'ores et déjà recueilli un avis favorable du Conseil d'État. Ce texte n'est pas concurrent de la loi sur les mobilités, il est concurrent des ordonnances. Nous ne remettons pas en cause le principe du recours à l'ordonnance, c'est une modalité constitutionnelle de législation qui est encadrée. nous sommes probablement nombreux dans cet hémicycle à avoir soutenu, au moins une fois, un gouvernement qui se proposait de légiférer par ordonnance. La question, c'est l'opportunité d'utiliser ce procédé sur ce sujet particulier. Ce qui est choquant, c'est de réformer le système ferroviaire par ordonnances. Nous sommes les représentants des territoires. Nous avons trop à dire sur ce sujet stratégique d'aménagement du territoire. Nous ne pouvons pas être privés de ce débat nationales de la mobilité ont exclu le sujet du ferroviaire au motif que des rapports importants étaient attendus. Et maintenant, il serait trop tard ? C'est la mission du Sénat de faire entendre la voix des territoires. Le Gouvernement ne peut pas se priver de ses contributions, vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, le débat doit porter ses fruits et nourrir la réforme. Il doit avoir lieu, et il s'engage ce soir, grâce au texte de Louis Nègre et d'Hervé Maurey. Sur le fond, les ordonnances gouvernementales semblent devoir ne proposer qu'une transposition sèche du droit européen.

Voici la principale divergence entre les ordonnances et notre texte : tandis que les rapports Borne et Spinetta préconisent une ouverture à la concurrence en pur, nous proposons des « packages territoriaux », des « lots ». Autrement dit, il ne faut pas mettre sur le marché les lignes les plus rentables que tout le monde voudra, sans contrepartie de desserte territoriale. Ce que propose le présent texte est de n'attribuer les lignes rentables qu'en contrepartie d'engagements d'exploitation et de desserte du réseau secondaire sur une zone géographique donnée. Nous sommes à l'heure où la logique comptable étouffe les territoires ruraux, à l'heure où, en brandissant une implacable calculette, on nous explique qu'il n'y a pas d'autre choix que de fermer des écoles et des classes, de fermer des services hospitaliers et des maternités, de fermer des trésoreries et des bureaux de poste, et même de diminuer le nombre de parlementaires Faisons le choix, pour une fois, de protéger sciemment certains services « non rentables », en les considérant comme des éléments structurants indispensables des territoires ruraux. Faisons ce choix avant que les lignes secondaires n'aient disparu Madame la ministre, entendez notre inquiétude. Nous connaissons bien, nous qui sommes élus ruraux, le sens du terme « redéploiement », qui ne signifie, dans nos campagnes, que fermetures et éloignement des services. Nous n'en pouvons plus ! Les électeurs perdent patience et confiance Cette réforme pose d'autres problèmes sur lesquels nous allons nous pencher : celui, bien évidemment, des modalités de transfert des salariés, celui de l'accès aux données de l'opérateur historique, celui du degré d'exigence en termes de normes environnementales, celui du transfert des gares et du matériel, celui de la dette chronique et croissante de SNCF Réseau. Mais le seul cap que nous devons avoir, c'est l'amélioration du service aux usagers, à l'occasion de ce qui doit être une impulsion nouvelle. Le groupe Union Centriste votera donc la proposition de loi Maurey-Nègre, qui est, pour une fois, un vrai texte d'aménagement du territoire. Je souhaite, pour conclure, citer notre auteur nivernais, Jules Renard, qui disait, au début du XX siècle : « Le train,

Je veux aussi saluer les objectifs qui ont guidé ce travail, qui sont les mêmes que les vôtres, madame la ministre : améliorer la qualité et réduire le coût du service, plaçant ainsi l'usager, le voyageur au coeur de nos préoccupations.

en contrepartie de la réalisation d'obligations de service public définies en fonction des besoins d'aménagement du territoire ». Une telle disposition répond aux préoccupations que j'ai pu moi-même, comme d'autres, exprimer dans cet hémicycle à plusieurs reprises. La desserte fine de nos territoires par le TGV ne doit pas être remise en cause. La logique purement financière ne doit pas se substituer à l'aménagement du territoire. Je le dis

Ce qui nous inquiète, c'est, bien sûr, le maillage de nos territoires par les trains régionaux qui relient les territoires les uns aux autres. Je pourrais citer l'exemple de la liaison Strasbourg-Saint-Dié,

et participe très souvent aux investissements de régénération. Il est donc important d'encadrer l'ouverture à la concurrence afin d'éviter que, là aussi, la logique financière ne domine. Vous avez affirmé que vous étiez opposée à cette fermeture des « petites lignes », une expression que vous n'aimez pas, vous

Il a également été reconnu comme étant le cinquième meilleur réseau du monde, derrière la Suisse, le Japon, Hong Kong et Singapour. Malgré cela, des défaillances sont régulièrement constatées, et les récents incidents nourrissent une appréciation mitigée des Français envers l'opérateur historique. Si la qualité du service doit être améliorée, l'ouverture à la concurrence constitue l'opportunité pour l'opérateur historique d'aller dans ce sens. Celle-ci est une obligation européenne depuis l'adoption du quatrième paquet ferroviaire, comme cela a été rappelé. Ce corpus de textes européens impose l'ouverture à la concurrence des TER et des trains d'équilibre du territoire dès le 3 décembre 2019. Pour les services commerciaux, c'est-à-dire les TGV, cette libéralisation devra être prévue par la loi à partir du 1 janvier 2019, pour une application effective à partir du 14 décembre 2020. La proposition de loi de notre collègue et président de commission Hervé Maurey et de l'ancien sénateur Louis Nègre, dont nous débutons l'examen ce soir, est le fruit de nombreuses auditions et consultations. Elle vise à mettre en oeuvre cette ouverture à la concurrence et à garantir son effectivité. Les Français regardent outre-Manche et aspirent à une concurrence différente de celle qui a été instaurée au Royaume-Uni, pays qui ne brille pas par son transport ferroviaire. Regardons plutôt chez nos voisins italiens, allemands ou suédois et voyons ce qui marche. Il faut s'y prendre tôt pour réussir cette transformation, mais les craintes sont nombreuses, les freins aussi. Le texte que nous abordons tend à lever les obstacles à une ouverture effective du transport ferroviaire à la concurrence, en ce qui concerne notamment l'accès des entreprises ferroviaires aux données nécessaires à la préparation des candidatures aux appels d'offres et à l'exploitation des services, sans oublier le transfert du personnel, la propriété des matériels roulants, l'accès aux ateliers de maintenance et aux gares. Je n'entrerai pas dans le détail des dispositions de cette proposition de loi, car cela a été fait avant moi. Je tiens néanmoins à rappeler la problématique de l'aménagement du territoire. Certes, certaines lignes sont rentables et d'autres le sont beaucoup moins. Mais nous devons veiller à toujours maintenir ces lignes, comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, même si elles sont déficitaires, pour ne pas abandonner le milieu rural. L'activité économique, la vitalité des territoires ruraux en dépendent. La desserte des territoires ruraux doit continuer à être effectuée. Dans le cas contraire, si les lignes étaient amenées à disparaître, certains départements verraient leur population décroître progressivement. l'amélioration des lignes existantes constitue un objectif, il n'est jamais question des projets de réouverture de ligne. Or ces projets doivent être encouragés par l'État. Dans mon département, la Haute-Savoie, la croissance démographique explose. Avec 820 000 habitants, la population haut-savoyarde a augmenté de plus de 20 % en moins de dix ans. Madame la ministre, je reparlerai d'un projet qui m'est cher, mais qui n'a toujours pas eu de réponse de votre part : la réouverture de la ligne du Tonkin ou RER Sud-Léman. Il s'agit d'un projet franco-suisse. La ligne ferroviaire d'Évian-les-Bains à Saint-Gingolph est le dernier maillon dans la boucle ferroviaire du lac Léman, en continuité du Léman Express, qui verra le jour en décembre 2019. SNCF Réseau a donné son feu vert à ce projet de réouverture aux voyageurs, qui permettra de désenclaver l'est du Chablais. de désenclaver l'est du Chablais. Il est soutenu par les collectivités françaises et suisses. La région a reconfirmé son engagement. Considérant l'importance de ce projet pour notre territoire, la réaffirmation des soutiens du côté français-

que nous portons avec Marion Lenne, députée du Chablais, mais également avec les élus français et suisses et les associations. Il est fondamental de penser à la mobilité du futur. Sur le plan écologique, soulignons aussi que, si le rail reste l'un des modes de transport les plus écologiques, les usagers s'en détournent aujourd'hui peu à peu en raison du coût élevé, des retards et, désormais, des grèves. Ils ont d'autres options à leur disposition : le transport par bus, le covoiturage en sont quelques-unes. La libéralisation me semble indispensable à la survie du transport ferroviaire de voyageurs, face à la concurrence exacerbée des autres modes de transport. Je voterai en faveur de cette proposition de loi. C'est pourquoi je souhaite à mon tour remercier notre collègue rapporteur, Jean-François Longeot, pour la qualité de son travail. Pour conclure, je rappellerai que supprimer le monopole de la SNCF ne signifie pas s'opposer à cette entreprise. Je tiens, au passage, à saluer l'investissement des femmes et des hommes qui y travaillent. L'arrivée de nouvelles entreprises ferroviaires sur le marché doit certes permettre l'émergence de nouveaux services, de meilleure qualité et à un moindre coût, mais elle doit aussi encourager l'opérateur historique à offrir des services plus performants. La parole

temps, je pense qu'on peut tous faire le constat que nous sommes aujourd'hui face à des impasses, qui sont d'autant plus complexes qu'on a trop tardé. Par exemple, quand le quatrième paquet ferroviaire a été adopté- cela ne date pas d'hier, puisque cela remonte à 2015 -, on aurait pu se préoccuper de préparer l'ouverture à la concurrence. On aurait pu aussi se préoccuper par le passé de traiter le modèle économique du système ferroviaire. Je rappelle que, jusqu'à présent, n'avait considéré que la dette du ferroviaire était un problème. Je rappelle aussi que le précédent gouvernement a même remis un rapport au Parlement expliquant que la dette n'était pas un problème. C'est pourquoi, aujourd'hui, le Gouvernement doit conduire une réforme globale, dont je redis qu'elle passe par un investissement massif

à leurs habitants et à leurs entreprises. Je voudrais également redire qu'il n'est pas question de régionaliser les lignes UIC 7 à 9.

Ces lignes recouvrent des réalités très différentes : certaines sont des capillaires fret- elles représentent 30 % à 40 % du trafic de fret ferroviaire et sont à ce titre essentielles

d'écrire le projet de loi qui pourra être débattu sur le fond à l'Assemblée nationale et dans votre assemblée. J'ai eu l'occasion d'indiquer aux organisations syndicales et aux représentants des entreprises et des régions

travers celui-ci, nous souhaitons porter une idée simple : la France ne peut pas être simplement l'exécutant zélé de la Commission européenne.

Les monopoles ont été brisés et les marchés ouverts à la concurrence sans qu'aucun bénéfice puisse être mis en exergue pour les usagers ou pour la société dans son entier. L'Europe du rail est encore un voeu pieux. Partout en Europe, ces recettes produisent la disparition de lignes, l'explosion des prix, la vétusté des installations et des trains, la disparition du fret et la diminution du nombre de cheminots. En Angleterre, les tarifs ont explosé. En Italie, l'ouverture à la concurrence s'est traduite par une multiplication des accidents. En France, l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire a conduit à une réduction de l'offre, à des infrastructures laissées à l'abandon et à une activité abandonnée,

48 000 morts par an. Pouvons-nous réellement continuer comme cela ? Nous estimons donc qu'il convient que la France propose à ses homologues européens, avant toute nouvelle législation en la matière,

Nous souhaitons également la réalisation d'un bilan carbone des politiques de libéralisation du transport ferroviaire. En effet, tout report sur la route a des conséquences désastreuses. Les transports sont l'un des secteurs les plus émissifs. Il s'agit donc d'un véritable levier pour donner du sens aux engagements européens en faveur du report modal et d'une baisse globale des émissions de gaz à effet de serre, conformément aux accords pris dans le cadre de la COP 21. Quel est l'avis de la commission ?

ce qui est contraire au principe de séparation des pouvoirs. Dès lors, notre commission n'a pu émettre qu'un avis défavorable. Quel est

Les émissions ont même augmenté de 0,9 % en 2015 en France, selon les derniers chiffres dont nous disposons. Pis, deux ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, les résultats sont décevants selon ces chiffres provisoires, publiés par le ministère de la transition écologique, en 2016, la France aurait émis 463 millions de tonnes de gaz à effet de serre, en hausse par rapport à 2015. Il nous semble dès lors qu'il est plus que temps que les pouvoirs publics interviennent et créent un cadre juridique qui permette de limiter ces émissions. Dans ce cadre, le développement du fret ferroviaire est un levier important. En effet, alors que le Grenelle de l'environnement souhaitait porter la part du fret non routier à 25 % à l'horizon de 2022, chaque année le fret ferroviaire perd des parts de marché. Aujourd'hui, il représente moins de 10 % du fret global. Alors que le réseau routier s'est largement développé en trente ans, le réseau ferroviaire, lui, a régressé. Cette situation est la conséquence directe des politiques de désengagement de l'État de ce secteur d'intérêt général. La politique de volume a été remplacée par la volonté de développer uniquement les autoroutes ferroviaires, au détriment de l'activité du wagon isolé. À l'inverse, nous proposons de longue date de déclarer le fret d'intérêt général. Nous l'avons encore proposé au Sénat en décembre dernier au travers d'une proposition de résolution.

La décision récente de la Commission européenne sur le cas italien crée ainsi un précédent bienvenu pour investir dans le rail sans risque de distorsion de concurrence. La France, qui a accueilli la COP 21, se doit d'être exemplaire dans ses politiques environnementales. Pour cela, il convient de déclarer le fret ferroviaire d'intérêt général. Quel

ou par des objectifs de part de marché, mais bien par des actions concrètes. Il faudrait notamment restaurer une concurrence plus loyale de la part du transport routier, ce qui passe notamment

des poids lourds qui transitent sur notre territoire au financement des infrastructures. Cela permettra d'avoir une concurrence plus équitable entre le rail et la route. Cela passe en outre par des investissements qui puissent garantir des sillons de qualité. C'est tout le travail qui a été fait dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures. Cela passe enfin par une politique de péages

est de mettre en place une politique de ferroutage, de mettre au gabarit européen certains tunnels par lesquels les conteneurs ne peuvent passer et de faire en sorte qu'on réhabilite les voies

Certes, le service n'était pas totalement performant, et l'usine ignorait parfois où se trouvait le wagon, mais, dans la très grande majorité des cas, il finissait par arriver. Il a fallu se battre à un certain moment pour le maintenir, puis il y a eu une seconde attaque, et ce service a disparu. Aujourd'hui, ces matières, qui sont dangereuses, sont transportées par camion : c'est une aberration une aberration ! En second lieu, dans le même département, une communauté de communes, devenue communauté d'agglomération, a réalisé une zone de développement économique qui est reliée à la voie ferrée. Les travaux de raccordement sont réalisés, et l'entreprise qui s'installerait là n'aurait qu'à faire rouler ses wagons et à terminer la voie ferrée jusqu'à ses bâtiments. Or, en une dizaine d'années,

nous souhaitons tracer les lignes d'une politique des transports permettant d'engager notre pays dans la voie du service public et de l'intérêt général. Dans ce cadre, comme nous l'avons déjà évoqué, la question du report modal de la route vers le rail semble centrale, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

ce simple exemple : les opérateurs du rail participent au financement des infrastructures par le paiement de redevances à SNCF Réseau. Il n'en est pas ainsi pour la route, dont l'usage, hors autoroute autoroute concédée, est purement gratuit et totalement financé par les pouvoirs publics. Cet amendement, reprenant une proposition que nous avons formulée dans la proposition de loi permettant la relance du secteur public ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique déposée en 2012, prévoir que toute opération de transport routier de marchandises doit aussi prendre en compte les coûts d'entretien des infrastructures, qui sont aujourd'hui supportés par les seules collectivités, et les coûts externes. Je précise que les coûts externes sont les coûts des effets négatifs du transport qui ne sont pas payés par les usagers eux-mêmes. Il en est ainsi des coûts du changement climatique, du coût de la pollution et de ses conséquences sanitaires, du bruit, de l'encombrement, autant d'éléments qu'il convient de prendre en compte dans la tarification des transports routiers. Dans le même sens, la Commission européenne estime qu'un se dégage parmi les scientifiques sur le fait que les coûts externes du transport peuvent être mesurés des approches axées sur les meilleures pratiques et que des chiffres sont prêts pour être utilisés

en faveur du fret ferroviaire, en intégrant les coûts externes du transport routier dans sa tarification. Cela permettrait également de lutter contre le dumping social, qui se traduit souvent par une sous-tarification du service. Quel est l'avis de la

M. Guillaume Gontard. Nous proposons un moratoire sur la fermeture des gares de triage, qui sont essentielles pour le maintien et le développement du fret ferroviaire, pilier de la transition écologique. On rappellera une nouvelle fois cet objectif d'intérêt général ainsi que les engagements de la France lors des accords de Paris. Comment comptons-nous mettre en oeuvre cette transition si nous laissons le fret ferroviaire perdre du terrain face au fret routier ? Le développement du fret est un outil indispensable pour diminuer la circulation massive des poids lourds et la pollution, ainsi que la gêne qu'elles engendrent. Ainsi, nous proposons un moratoire sur la fermeture des gares de triage, dont la résorption est un non-sens écologique. Nous étions presque unanimes sur ce point lors de l'examen de la proposition de résolution de notre groupe voilà à peine trois mois. Nous vous invitons donc, chers collègues, à voter cet amendement, en cohérence avec nos positions antérieures.

est à M. Fabien Gay. Par cet amendement simple, nous souhaitons affirmer une position de principe, qui tend à être mise à mal par les réformes successives. successives. Nous estimons que le réseau ferré national, construit principalement grâce à l'impôt de nos concitoyens, doit être exclusivement détenu par la puissance publique, afin d'affirmer non seulement sa cohérence et sa pertinence, son unicité, qui garantit l'accès au service public des transports, donc au droit de toutes et tous à la mobilité. Nous ne partageons évidemment pas l'idée confortée par le rapport Spinetta qu'il faudrait se dessaisir des petites lignes, sacrifiant ainsi près de 9 000 kilomètres de réseau.

Le nouveau pacte ferroviaire, comme cette proposition de loi qui organise la concurrence pour les TER, Intercités et autres TGV, risque, sous couvert de mise en concurrence, de renforcer ce mouvement. Les régions se voient attribuer, réforme après réforme, des compétences nouvelles, y compris par cette proposition de loi, qui prévoit de confier aux régions la propriété du matériel roulant et des ateliers de maintenance. Elles ne peuvent assumer un tel transfert de charge sans les moyens qui vont avec. Le succès de la décentralisation des TER s'est faite au prix que cette charge devienne le premier poste de budget des régions. Le succès a tenu également aux relations tripartites entre l'État, les régions et la SNCF. La multiplication des opérateurs altérera la cohérence globale de l'offre interrégionale et renforcera les fractures territoriales.

Cette situation est très étroitement liée aux injonctions de la directive de 1991, à savoir inviter les États à réduire l'endettement des compagnies ferroviaires. Dès cette période, l'État français, à l'image de ce qui s'est opéré en Allemagne, aurait pu faire le choix de reprendre l'ensemble de la dette à son compte. Malheureusement, ce n'est pas la voie qui a été choisie.

Nous proposons donc, à l'instar du principal syndicat du secteur, la création d'une structure de défaisance, caisse d'amortissement de la dette ferroviaire qui serait financée par le produit des concessions autoroutières, dont nous préconisons par ailleurs la nationalisation. Le seul obstacle à la reprise de la dette par l'État est le respect des règles de Maastricht concernant le déficit public. Il faut pourtant pouvoir s'en affranchir pour le bien de la Nation et des usagers du service public ferroviaire. en effet que les intérêts de la dette, qui représentent chaque année 1,7 milliard d'euros, seraient bien plus utiles au financement des infrastructures qu'à celui des banques.

et les solutions qui pourraient être mises en oeuvre, notamment la création d'une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire. Ce rapport a bien été rendu en 2016, mais il n'a absolument pas résolu la question, la renvoyant au gouvernement suivant.

l'avis du Gouvernement ? Je vous confirme que le Gouvernement a souhaité engager une réforme globale, qui vise notamment à remettre à l'équilibre la trajectoire financière du secteur ferroviaire. Dans ce cadre, comme le Premier ministre a eu l'occasion de l'indiquer, le Gouvernement

dans d'autres sphères, que la dette serait celle des cheminots. C'est un point heureux de cette discussion. La dette est surtout le résultat des injonctions contradictoires auxquelles